La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 6 juillet 2017 a été publié sur le site internet du Sénat.

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, c'est avec tristesse que nous avons appris hier le décès de notre ancien collègue Robert-Paul Vigouroux, qui fut sénateur des Bouches-du-Rhône de 1989 à 1998. Neurochirurgien au talent mondialement reconnu, il adhéra à la SFIO en 1964 et s'engagea dans la vie politique marseillaise aux côtés de Gaston Defferre. Il fut élu conseiller général en 1967 et entra au conseil municipal de Marseille en 1971. Devenu maire de Marseille au décès de Gaston Defferre, en 1986, il fut brillamment réélu à l'occasion des élections municipales de 1989. Il fut, à la tête de la cité phocéenne, l'initiateur de plusieurs grands projets d'aménagement, notamment du vaste quartier Euroméditerranée. Élu sénateur en 1989, il se rattacha au groupe socialiste, puis au groupe du RDSE. Il fut membre de la commission des affaires étrangères, puis de la commission des lois. Au nom du Sénat, je veux assurer sa famille et ses proches, ainsi

Je vous remercie,

de recueillement en sa mémoire. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

nous vous accueillons avec plaisir, pour cette première prise de parole en séance publique au Sénat.

monsieur le président et rapporteur de la commission des lois, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, conformément à l'engagement pris devant les Français par le Président de la République, vous êtes aujourd'hui saisis d'une réforme très attendue, je crois, par nos concitoyens, et dont l'ambition est de rétablir la confiance dans l'action publique.

l'honneur de présenter devant vous, au nom du Gouvernement, ces deux textes. La transparence, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent une exigence sociale, politique et éthique fondamentale. Le respect de cette exigence a toujours constitué le fondement de la confiance que les citoyens éprouvent à l'égard de leurs gouvernants comme de tous ceux qui concourent à l'exercice Est-il nécessaire de rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame, en son article XV, que « la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration » Ce principe de confiance est donc ancré dans notre histoire depuis longtemps et, ces dernières années, beaucoup a été fait pour mieux répondre à des exigences nouvelles. Plusieurs textes ont été adoptés sur ces sujets. Je me contenterai de les énumérer brièvement : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la loi la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui a institué un procureur de la République financier, la loi du 20 avril 2016, qui a renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires plus récemment, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a notamment créé l'Agence française anticorruption.

beaucoup reste encore à faire pour restaurer cette confiance, nécessaire dans une démocratie, entre les citoyens et leurs représentants. Je souhaite le dire d'emblée et être très claire sur les intentions du Gouvernement il n'est aucunement question ici de stigmatiser le comportement de l'ensemble des élus locaux et nationaux, dont l'engagement exemplaire doit être sans cesse rappelé.

Je suis convaincue que le rétablissement de cette confiance permettra aux citoyens d'apprécier l'engagement des élus sous son meilleur jour et leur volonté d'agir efficacement dans le sens de l'intérêt général sans compter leur temps ni leurs efforts. Je sais cela suffisamment pour pouvoir l'affirmer ici avec force. C'est précisément pour cela que nous avons collectivement besoin d'un choc de confiance.

Par cette réforme, le Gouvernement entend apporter une réponse globale, fondatrice, en proscrivant définitivement certaines pratiques, mais également en renforçant la transparence et le pluralisme de la vie politique. Tout en édictant de nouvelles règles qui renforcent les garanties de probité et d'intégrité des élus et la prévention des conflits d'intérêts,

Elle répond à quelques principes simples : sanctionner plus sévèrement ceux qui manquent à la probité et éviter les conflits d'intérêts ; mettre fin à des pratiques qui ne sont plus acceptées par les citoyens renforcer les contrôles sur les comptes des partis, tout en leur offrant, ainsi qu'aux candidats, un accès plus facile au financement, un moyen de garantir la réalité du pluralisme. J'évoquais la prise de conscience collective qui nous conduit à cette réforme et je voudrais rendre hommage à votre commission des lois, de même qu'à son président-rapporteur, M. Philippe Bas, qui a montré ces derniers jours sa volonté de s'inscrire résolument dans cet esprit. Les travaux de votre commission des lois, comme ceux d'ailleurs de la commission des finances et de son rapporteur pour avis, Albéric de Montgolfier, ont été marqués par une démarche collective et par une grande richesse des débats, qui ne manqueront pas de caractériser également, j'en suis sûre, les échanges dans cet hémicycle.

elle s'attache à l'exercice du mandat parlementaire, elle renforce les règles de probité des acteurs, et elle conduit à une refonte des règles de financement de la vie politique.

et parce qu'ils représentent le peuple, parce qu'ils incarnent la souveraineté nationale, les parlementaires sont tenus à un devoir d'exemplarité particulièrement exigeant. Vous devez pouvoir légiférer et contrôler l'action du Gouvernement en toute indépendance, sans subir en aucune manière le jeu des puissances ou des. Je sais combien vous êtes attachés à cette indépendance.

Un renvoi au règlement des assemblées pour la mise en oeuvre des dispositions a ainsi été prévu chaque fois que nécessaire, dans la limite du champ de compétence défini par le Conseil constitutionnel, à savoir l'organisation ou le fonctionnement des assemblées, la procédure législative et le contrôle de l'action du Gouvernement. Votre commission a parfois adapté les dispositifs en prévoyant la compétence du bureau du Sénat ; le Gouvernement comprend les raisons qui peuvent dicter ce choix. Je précise en outre que, chaque fois que cela se justifiait, les mesures applicables aux parlementaires nationaux ont été étendues aux représentants français au Parlement européen.

de nouveaux cas d'inéligibilité et d'incompatibilité sont créés. En premier lieu, les parlementaires dans l'incapacité de justifier qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales ne pourront plus rester en fonction. Saisi par le bureau de l'assemblée, le Conseil constitutionnel pourra prononcer la démission d'office du parlementaire. En second lieu, les incompatibilités relatives à l'activité de conseil sont renforcées et étendues. À l'heure actuelle, seule l'impossibilité pour un parlementaire de commencer, pendant son mandat, une activité de conseil existe. Cette interdiction ne s'applique d'ailleurs pas aux professions libérales réglementées, comme la profession d'avocat. Cette disposition est apparue très insuffisante en raison des risques de conflits d'intérêts liés à ce type d'activité. Ce dispositif est donc complété selon trois axes un parlementaire ne pourra commencer à exercer de telles activités pendant son mandat et devra cesser celles qui ont débuté au cours des douze mois précédant le début de son mandat. La dérogation qui s'applique pour les professions réglementées est par ailleurs supprimée. les fonctions de direction exercées dans une société de conseil sont désormais prises en compte. Enfin, le contrôle par un parlementaire d'une société de conseil est également visé. un parlementaire qui détient une société de conseil peut être influencé par les intérêts de ses clients, comme s'il en était le dirigeant. Actuellement, le code électoral ne prévoit rien ; le projet de loi y remédie. Le dispositif proposé par le Gouvernement en matière d'encadrement des activités de conseil assure une conciliation entre les objectifs d'intérêt général visés par le texte, tels que l'indépendance des élus ou la prévention des risques de conflits d'intérêts, et et d'autres droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier la liberté d'entreprendre reconnue au parlementaire comme à tout citoyen. Les dispositions prévues devraient permettre d'éviter les écueils constitutionnels mis en évidence par la décision du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013, qui avait censuré une interdiction trop générale.

Le choix assumé du Gouvernement est de retenir une définition de la notion de conflit d'intérêts moins englobante que celle qui figure dans les lois du 11 octobre 2013 et du 20 avril 2016. Ce choix est justifié par le souci de ne pas mettre les parlementaires exerçant d'autres responsabilités, notamment électives, les conduisant à assumer un autre intérêt public, par exemple local, un autre intérêt public, par exemple local, dans l'impossibilité récurrente de participer aux travaux du Parlement. Il reviendra à chaque assemblée de préciser les règles internes de prévention et de traitement de ces situations de conflits d'intérêts. Troisième aspect, dans un souci de transparence concernant les frais engagés par les parlementaires dans l'exercice de leur mandat, le projet du Gouvernement a prévu que l'indemnité représentative de frais de mandat, l'IRFM, soit remplacée par un remboursement de ces frais, sur une base réelle et sur présentation de justificatifs. La commission des lois a adopté un nouveau dispositif dont nous débattrons, le Gouvernement étant attaché à quelques principes simples et lisibles sur ce sujet il appartient aux assemblées de définir les conditions et les plafonds de remboursement des frais de mandats ; les frais doivent naturellement être réellement exposés et faire l'objet de justificatifs ; ils doivent faire l'objet de remboursements et non d'une indemnisation. Nous

ouvert à la discussion sur ce point, mais estime que ce débat doit avoir lieu en loi de finances, ce qui est naturel pour un dispositif de nature budgétaire.

Premièrement, les obligations de transparence pesant sur le Président de la République sont renforcées. Chaque citoyen pourra juger de l'évolution de son patrimoine entre le début et la fin de son mandat, au regard de l'avis publié par la Haute

crime et pour une série d'infractions à la probité comme la corruption, le détournement de fonds publics ou encore la fraude électorale ou fiscale, dans le respect du principe de nécessité des peines garanti par l'article VIII de la Déclaration de 1789 1789 et du principe d'individualisation des peines, qui en découle. Seront ainsi écartées des fonctions électives les personnes qui ont démontré qu'elles ne remplissent plus les conditions de moralité essentielles à l'exercice d'un mandat électif.

aux parlementaires et aux titulaires de fonctions exécutives locales d'employer des membres de leur famille proche comme collaborateurs. Cette pratique acceptée hier ne l'est plus aujourd'hui. Cette interdiction est déjà prévue, pour ce qui concerne les collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement, par le décret du 14 juin 2017, conformément au principe de séparation des pouvoirs. Des dispositions

Les partis politiques dépendent très largement du financement public. Néanmoins, les règles qui s'appliquent à eux n'offrent pas toutes les garanties contre les abus ou les dérives. Ces règles sont par ailleurs peu favorables au renouvellement de la vie politique et au pluralisme. Il est donc proposé, tout d'abord, tout d'abord, de renforcer le contrôle des comptes des partis politiques et des campagnes électorales, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la Constitution, selon lequel « les partis et groupements politiques [ ...] se forment et exercent leur activité librement. le mandataire financier du parti recueillera l'ensemble des ressources reçues par ce dernier et non plus seulement les dons. Les partis politiques devront tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables. Cette comptabilité devra inclure les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement, afin de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de disposer d'un périmètre de contrôle consolidé. La question se pose de savoir si ces obligations doivent être ou non étendues à tous les partis, même à ceux qui ne relèvent pas de la loi du 11 mars 1988. Votre commission des lois l'a souhaité, pour y intégrer les micropartis. Cette extension pose certaines difficultés, que nous évoquerons lors de l'examen de l'article concerné.

Une interdiction des prêts des personnes morales, y compris de droit étranger, à l'exception des partis et des établissements de crédit européens est également posée. posée. Toutefois, en contrepartie, l'accès au financement par les candidats et partis politiques sera amélioré grâce à la création d'un médiateur du crédit, que votre commission a a souhaité désigner sous un autre titre. Nous y reviendrons. Enfin, le Gouvernement souhaite la création d'une structure pérenne de financement, la banque de la démocratie, afin de remédier aux carences du financement bancaire privé. Cette banque pourra se constituer sous la forme juridique d'un établissement doté de la personnalité morale, être adossée à un établissement de crédit existant ou prendre la forme d'un mécanisme de financement spécifique. Une mission va être confiée en ce sens à l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration, pour étudier les conditions de mise en place de cette structure. Il semblerait que nous ayons là une divergence avec votre commission des lois.

en lui apportant, je le répète, un surcroît de transparence, de justice et d'éthique. Elles sont à la fois ambitieuses et équilibrées ambitieuses, parce qu'elles s'attaquent aux vraies questions que se posent nos concitoyens depuis plusieurs années et singulièrement au cours des derniers mois de poser des interdits, mais aussi de consolider le pluralisme politique dans notre pays, la transparence de notre vie démocratique et, ainsi, la confiance de nos concitoyens dans les institutions et leurs représentants. Comme vous le savez, ces mesures seront complétées par la réforme constitutionnelle annoncée par le Président de la République dans son discours au Congrès du Parlement, le 3 juillet dernier. Il s'agit donc ici du premier acte, inaugural, essentiel, de cette volonté de rétablir le lien de confiance entre les Français et leurs élus.

Assemblée. Il souhaite que cette réforme volontariste et souhaitée par les Français soit à la hauteur de leur attente. Le président Bas s'est réjoui

Madame la garde des sceaux, c'est un honneur pour le Sénat d'être saisi en premier de ces projets, annoncés comme très importants par le Président de la République et le Gouvernement. Le Sénat est naturellement disponible pour aller de l'avant dans ces domaines.

car il sait bien que son apport peut être repoussé par les pouvoirs alignés, qui sont autour du Président de la République comme la limaille de fer dans un champ magnétique en présence d'un aimant.

la séparation des pouvoirs et l'autonomie des deux assemblées, comme l'exige notre Constitution, dans l'intérêt même de la démocratie. À cet égard, nous défendrons l'égalité de traitement des parlementaires et des membres du Gouvernement ou des responsables exécutifs. exécutifs. Bien sûr, nous défendrons aussi notre propre travail, car, au fil des années, sous l'impulsion notamment de notre président, Gérard Larcher, nous avons pris de l'avance dans nombre des domaines qui font l'objet des dispositions des deux textes présentés par le Gouvernement. Ainsi, en ce qui concerne les règles applicables à l'indemnité représentative de frais de mandat, nous avons tous dans notre poche le petit guide vert qui précise ce que nous avons le droit de faire et ce qui nous est interdit, le bureau

été par Jean-Jacques Hyest. Nous avons réglementé les emplois familiaux, pour en restreindre l'importance. Nous avons posé des règles pour l'accès au Sénat des représentants des et

de législation. C'est dire que le Sénat a de multiples raisons de s'engager dans la discussion de ces textes l'esprit serein

pas un. C'est d'ailleurs heureux, car des centaines de milliers de Français peuvent avoir un litige tout à fait légitime avec l'administration fiscale sans pour autant être des fraudeurs. Nous savons tous à quel point le code général des impôts est complexe et peut donner lieu à des interprétations contradictoires, si bien que vous avez limité cette exigence à l'obligation, pour le contribuable devenu parlementaire,

Nous avons traité de la question des intérêts, en demandant que les règles de déport appliquées aux parlementaires le soient aussi, en conseil des ministres, aux membres du Gouvernement. Nous avons souhaité que les frais de mandat soient pris en charge par les assemblées sur la base de justificatifs, nous inspirant du système anglais, qui passe pour le plus rigoureux au monde. Ce faisant, nous avons essayé d'éviter l'excessive rigidité qui caractérisait votre texte. Nous avons également voulu que les collaborateurs collaborateurs appartenant à la famille d'un parlementaire ne soient pas injustement pénalisés et qu'on leur laisse le temps de se retourner, de sorte qu'ils ne soient pas moins bien traités que n'importe quel salarié de France qui perd son emploi. Cela me paraît tout de même être la moindre des choses. Nous proposons que les communes rurales, qui, avec les départements et les régions, ont perdu 9,6 milliards d'euros de dotations en trois ans, puissent continuer à bénéficier de fonds de l'État pour financer des projets signalés par les parlementaires, avec toutes les garanties de transparence voulues. Nous avions d'ailleurs déjà posé des règles en ce sens. Nous souhaitons que cette dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements voie le jour, en évitant tous les abus auxquels donnaient lieu les financements d'associations qui, parfois, étaient de simples officines politiques. Enfin, nous ne voulons pas

ce que vous voulez en faire, ni quelle serait sa configuration. Ce n'est pas acceptable ! L'article 38 de la Constitution exige que les modalités et les conditions

! Quant à la loi, elle ne crée pas la morale. Elle peut simplement créer des règles pour ceux qui ne la respectent pas spontanément et pour faire évoluer les pratiques. Une loi est-elle de nature à rétablir la confiance ?

La confiance reviendra quand le chômage reculera, comme en Allemagne et au Royaume-Uni, quand le pouvoir d'achat progressera, quand la sécurité des personnes et des biens sera assurée, quand le terrorisme

il nous a paru plus exact de qualifier ces textes de projet de loi organique et de projet de loi « relatifs à la régulation de la vie publique ». J'espère que cette sobriété ne vous choquera pas.

des dispositions des deux projets de loi que nous examinons aujourd'hui concernant, d'une part, la suppression de la dotation d'action parlementaire, et, d'autre part, l'habilitation qui serait donnée au Gouvernement pour créer un dispositif souvent présenté comme la « banque de la démocratie Le Gouvernement avance tout d'abord des motifs juridiques pour justifier la suppression de la « dotation d'action parlementaire »- c'est le terme que nous préférons au Sénat -, en évoquant tantôt un « contournement », tantôt une pratique « contraire » à l'article 40 de la Constitution,

Le Gouvernement met aussi en avant un risque de clientélisme. Cependant, si ces risques ont sans doute été réels par le passé, la transparence est, depuis 2013, totale. l'initiative du Sénat, les deux assemblées publient désormais elles-mêmes, sous forme de données ouvertes, la liste des subventions. Cette publicité est supérieure à celle de nombre de subventions versées par les services de l'État Le Gouvernement annonce aussi l'économie de 6 emplois d'administration centrale, ce qui n'est pas extraordinaire, d'autant que ces effectifs seront maintenus pour gérer la réserve dite « ministérielle ». Comme vous le savez, la dématérialisation des procédures avait été engagée et l'on pouvait en attendre une réduction sensible des coûts administratifs. Enfin, le Gouvernement évoque le respect de certains critères « normés alors que l'administration nous a confirmé que les critères de recevabilité des demandes de subvention ne se distinguaient pas de ceux qui sont applicables aux subventions de l'État pour des projets d'investissement. je rappelle que la dotation d'action parlementaire correspond à seulement 0,03 % des crédits du budget de l'État, soit 147 millions d'euros, dont un peu plus de 56 millions d'euros pour le Sénat, consacrés à plus de 80 % à l'investissement des collectivités territoriales. Elle apporte donc à l'investissement local un soutien qui n'est pas seulement symbolique dans le contexte actuel de baisse des dotations et subventions de l'État aux collectivités territoriales. Elle irrigue également le tissu associatif

lycées français, irrigation culturelle des territoires, travaux sur les bâtiments religieux des petites communes, opérations en faveur des commerces de proximité, développement du tourisme, actions éducatives dans l'enseignement scolaire, etc.

Nous proposons donc, en lien avec la commission des lois, d'inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements. Nous proposons également d'améliorer la transparence de la réserve ministérielle en imposant sa publication par la loi, en format ouvert, en, sachant qu'elle aurait vocation à disparaître si la dotation pour les communes n'était pas adoptée. Au-delà de l'investissement local, j'attends du Gouvernement, madame la garde des sceaux, qu'il nous précise ses intentions pour les programmes qui bénéficiaient de manière récurrente de la réserve parlementaire,

comme vous le savez, le dispositif qui devait initialement figurer dans le projet de loi a été retiré à la suite de l'avis du Conseil d'État, qui l'a estimé trop lacunaire. Il a donc été remplacé par une demande d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance. L'accès au crédit bancaire constitue évidemment un enjeu fondamental pour la démocratie, afin de garantir, comme le rappelait M. le rapporteur à l'instant, que l'article 4 de la Constitution est bien respecté concernant « les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation », et pour éviter le risque d'un financement opportun opportun des campagnes et des partis. Cependant, la demande d'habilitation qui nous est soumise, volontairement très large, ne repose sur aucune étude préalable des besoins et des mesures nécessaires pour y répondre.

conduisant à analyser avant de légiférer, donc de supprimer cet article. C'est ce qu'a fait la commission des finances, à l'unanimité. La parole est à M.

sur les sujets de financement, de transparence et de moralisation de la vie politique, depuis la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et les lois présentées par les précurseurs en la matière que furent Michel Rocard et Alain Juppé, jusqu'à la dernière loi du 11 octobre 2013,

L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ce qui ce serait matériellement impossible.

pour ce qui concerne les indemnités parlementaires, notre commission a pris une décision qui n'est pas sans intérêt ni sans effet. Et je pense que nous avons eu raison. Comme tout le monde le sait, les parlementaires

vice-présidence ou présidence du Sénat ... Nous proposons que ces indemnités-là, qui sont liées à l'indemnité parlementaire, soient fiscalisées, en toute transparence.

Cette ouverture de nos hémicycles va dans le bon sens et prouve notre volonté de coconstruire le débat en toute transparence. Au regard des nombreuses propositions formulées, des votes et des contributions déposés sur la plateforme, je suis sûre que cette consultation constituera une vraie réussite. ne jamais légiférer dans la précipitation, cela signifie ne pas mettre de côté certains points essentiels. Aussi, nous regrettons que les projets de loi traitent si peu des élus locaux. sont visés par le biais de nouveaux devoirs, nous aurions souhaité leur accorder de nouveaux droits. La question récurrente de la formation des élus locaux me semble, en effet, prégnante. Un élu mieux formé est un élu qui prévient mieux les conflits d'intérêts. Enfin, le renouvellement en profondeur des représentants nationaux,

Alors même que le Gouvernement prône la négociation collective, garante d'un droit du travail à la fois plus respectueux des salariés et plus adapté aux enjeux actuels, les collaborateurs parlementaires peuvent-ils en être exclus ?

Je tiens à remercier tout particulièrement le président de la commission des lois, Philippe Bas, qui a reçu toutes les parties prenantes de ce dossier complexe. Je remercie également la vice-présidente du Sénat, Françoise Cartron, qui préside l'Association de gestion des assistants de sénateurs, sorte entre le marteau et l'enclume, elle est gardienne des exigences sénatoriales, tout en étant soucieuse de ménager la dignité et la reconnaissance des collaborateurs, dont elle sait le grand travail.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ces projets de loi correspondent à un engagement pris par le Président de la République. Il est naturel que nous les examinions à l'aune de l'ouverture d'une nouvelle période de la vie publique.

Il me semble préférable de nous montrer lucides quant aux interrogations et aux critiques qui se développent dans notre société.

cette préoccupation, et parfois cette tentation critique, et d'avoir la force de caractère de prendre, comme le Gouvernement nous y incite, un certain nombre de dispositions. Je voudrais aussi dire,

d'une part, d'inéligibilités supplémentaires à la suite de condamnations pénales pour des faits contraires à la probité dans la gestion de ressources publiques,

collègue et ami, le président du comité de déontologie parlementaire qui me contredira. En revanche, la limitation des activités de conseil

qui a beaucoup compté dans l'écriture de la Constitution, avait un grand respect pour le parlementarisme britannique, dont il reste ici quelque chose

nous nous demandons si l'idée, au départ « vertueuse », comme l'on dit trop souvent, de supprimer ce lien direct ne s'est pas transformée en « fric-frac budgétaire

du statut de parti politique, ou plutôt la réalité de l'étiquette de parti politique, afin de bénéficier des moyens du financement public. Madame la garde

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, les textes que nous examinons aujourd'hui visent à répondre à la défiance de nos concitoyens seulement de certains comportements de femmes et d'hommes politiques, mais aussi des vases communicants entre fonctions électives ou ministérielles, fonction publique et postes et intérêts privés.

Cette situation est insupportable, tant pour nos concitoyennes et nos concitoyens que pour la grande majorité des élus qui ont à coeur le débat politique et la défense de l'intérêt de leurs administrés. Le nouveau chef de l'État a très vite annoncé sa volonté de présenter un projet de loi sur la « moralisation de la vie publique », rapidement devenu un projet de loi relatif à la « confiance dans la vie démocratique » pour finalement viser à rétablir « la confiance dans l'action publique ». Le président Bas nous propose, quant à lui, de « réguler » la vie publique. Cette diversité sémantique provient, à mon avis, d'une difficulté à délimiter le champ d'intervention du législateur. Quelle est la source de la perte de confiance évidente de la population dans ceux qui font la politique, membres du Gouvernement et élus, en particulier parlementaires ? Comment ne pas constater que le le nouveau pouvoir fait déjà face un rejet dans l'opinion, notamment s'agissant des ordonnances qui s'attaquent au code du travail, alors même qu'une victoire importante aux élections législatives aurait dû s'accompagner d'une popularité inédite la raison de cette perte de confiance ne provient pas d'une vision désenchantée de l'exercice du pouvoir, mais plutôt d'un doute profond sur l'utilité du vote pour obtenir les changements attendus. Absolument

depuis des décennies, c'est une vie meilleure, c'est le retour du plein emploi, ce sont des conditions de logement et de soins décents, ce sont des études gratuites et de qualité, ce sont des retraites permettant de vivre dignement, c'est une lutte résolue, efficace, pour une transition écologique échappant aux industriels et financiers. Ce sont l'absence de résultats et les promesses non tenues qui exaspèrent nos concitoyens. Ceux qui « ne sont rien », ceux qui n'ont pas grand-chose, ne supportent plus l'image de certains qui réussissent en violant la loi, en profitant de la situation acquise à travers leur vote.

Le dernier épisode des élections législatives est frappant : Emmanuel Macron et son gouvernement ont obtenu une large majorité à l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont minoritaires dans le pays, comme l'a illustré le vote de confiance à l'Assemblée nationale. L'opposition est donc totalement minorée par le rouleau compresseur de la VRépublique. Exactement ! Pourtant, le Président de la République, élu par un vote nécessaire face à Marine Le Pen et non par un vote d'adhésion, entend appliquer son programme à la lettre, armé des prérogatives exceptionnelles que lui accorde la Constitution de 1958, sans tenir compte le moins du monde de la relativité de son élection. Bien au contraire,

Irriguer la démocratie demande de casser la verticalité rigide qu'impose le nouveau pouvoir alors que le mouvement En Marche, qui se voulait révolutionnaire, me semble-t-il, visait à privilégier l'horizontalité. Comme trop souvent, on annonce des choses et on fait le contraire une fois élu. C'est de cela que le peuple a assez. Instaurer la proportionnelle intégrale et non un saupoudrage est une exigence pour rétablir la confiance. Le mode de scrutin actuel apparaît de plus en plus comme un miroir déformant et déformé de la volonté populaire. Il y a danger. Persister dans cette voie peut conduire à une remise en cause de l'institution parlementaire elle-même. Redonner dans le même temps ses pouvoirs au Parlement doit être une priorité : fin du 49-3, droit d'amendement pleinement restauré, en particulier en matière budgétaire, et pouvoir de contrôle accru sont des exigences. Comment redonner confiance au peuple dans son Parlement si les pouvoirs de ce dernier s'amenuisent en peau de chagrin ? Les sujets sont vastes, comme celui, par exemple, d'une justice au service de tous, accessible aux plus faibles et à l'indépendance confortée pour affronter les dérives constatées au sein du pouvoir politique. Le fonctionnement de la haute administration et ses relations avec le pouvoir politique doivent aussi être profondément modifiés, et les allers et retours entre ces deux mondes interdits. Que dire des excès du CAC 40, de l'explosion des fortunes, des profits indécents gagnés sur des vies asservies et parfois brisées, comme chez Whirlpool et GM&S ? La répartition des richesses est une clé essentielle du retour de la confiance dans notre système politique. comment moraliser et rétablir la confiance sans s'attaquer aux liens frappants entre médias, pouvoir politique et finance ? Qui n'a pas constaté, durant la dernière campagne présidentielle, l'influence de certaines chaînes d'information, tombées peu de temps auparavant aux mains d'hommes d'affaires comme MM. Drahi et Bolloré, qui avaient choisi leur camp et le défendaient bec et ongles. C'est vrai ! Comment ne pas noter également la proximité des instituts de sondage avec les allées du pouvoir ou de la bourse, voire des deux ? Le texte dont nous allons débattre peut apparaître utile pour poser quelques rustines sur un pneumatique au bord de l'explosion. Interdire les emplois familiaux, remettre en cause les réserves parlementaire et ministérielle, s'interroger sur les moyens de fonctionnement des élus, améliorer encore le tracé des financements des partis politiques et des campagnes électorales : ces mesures constituent parfois des évidences et toujours des progrès incontestables. Au cours de la discussion, nous apporterons notre soutien à de telles dispositions améliorées de façon souvent pertinente par le président et rapporteur de la commission des lois.

statut des collaboratrices et collaborateurs parlementaires, pour répondre enfin aux préoccupations très vives qui s'expriment, particulièrement au sein de notre assemblée, à quelques semaines du scrutin sénatorial.

Un aller et retour démocratique sur un tel sujet aurait sans doute été profitable. Vous n'en avez plus voulu, madame la garde des sceaux, ce qui me semble très dommageable. Mes chers collègues, un grand quotidien a produit un dossier sur la montée en puissance du secteur privé dans nos sociétés occidentales, tout particulièrement en France, vieux pays de mixité de l'économie, des intérêts privés, en un mot de l'argent,

que nous divergeons avec les partisans, parfois béats, de ces projets de loi. Le poison de l'argent distillé dans la vie politique ne peut être régulé, il doit être combattu, il doit être éradiqué. Pour reprendre les mots utilisés par le Premier ministre sur un autre thème, nous estimons nécessaire de « désintoxiquer » notre société de la finance, de l'argent facile, de l'argent qui corrompt. Pour notre part, trois siècles plus tard, nous serons guidés par Montesquieu, Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintiennent ou se soutiennent. Les forces des lois dans l'un, le bras du prince toujours levé dans l'autre [ ...]. Mais, dans un État populaire, il faut un ressort de plus, qui est la VERTU ». Citer

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, qu'il soit urgent de se préoccuper de la défiance des Français envers les institutions et le personnel politique est une évidence. Nul besoin de sondages, d'ailleurs dénués de toute rigueur scientifique, pour s'en convaincre. Il suffit de regarder les résultats des dernières élections : Emmanuel Macron aura été élu par seulement 43,6 % des électeurs inscrits, l'abstention et les votes blancs ou nuls atteignant, quant à eux, 34 % des inscrits. Le désintérêt pour les législatives a été encore plus grand : au second tour, l'abstention, plus les blancs et nuls, atteignaient 62,3 % du jamais vu pour une consultation de cette importance. Ce qui signifie donc que 32,8 % seulement des électeurs inscrits ont choisi leur candidat, soit un score moyen de l'ordre de 20 % pour les heureux élus. Merveilleux système qui transforme une poignée d'électeurs en majorité écrasante

affermira « les fondements du contrat social ». Les comportements indélicats, parfois clairement délictueux, d'un certain nombre d'élus ou d'administrateurs, s'ils n'arrangent évidemment pas les choses, ne sont pas l'explication fondamentale de la décrédibilisation de l'action publique et de ses acteurs. Comme la loi d'octobre 2013, née de la panique de l'Olympe face à « l'affaire Cahuzac », cette loi d'exorcisme n'a pas plus de chance de rétablir «la confiance dans l'action publique » que de mieux « réguler la vie publique ». Elle la compliquera seulement Destinée à faire oublier « l'affaire Fillon » et celles qui l'ont suivie, touchant, cette fois, la nouvelle majorité, elle n'est pas une réponse à cette sécession civique. Et ce d'autant moins qu'elle n'a plus grand-chose à voir avec l'intention première de son initiateur, François Bayrou, qui, lui, voulait « lutter contre l'influence des intérêts industriels et financiers dans la vie politique ». L'origine sécession, sur fond de langueur économique depuis 2008, de crainte de déclassement pour les classes moyennes, ou de précarisation pour les plus exposés, c'est le verrouillage du système politique, le constat que changer la tête de l'État ne revenait qu'à perpétuer la même politique particulièrement efficace. On comprend que ce système, dépourvu de perspectives, finisse par lasser et engendrer ce qui ressemble de plus en plus à des « émeutes électorales » aux effets imprévisibles. Réservant l'analyse du détail des projets de loi pour l'examen des articles, vous me permettrez de revenir sur les raisons de cette sécession civique et sur la fonction des boucs émissaires en post-démocratie libérale. Custine définissait le régime tsariste comme une « monarchie absolue, tempérée par l'assassinat ». Je dirais de la V République néolibérale qu'elle est une république oligarchique- oligarchie de la finance et de l'héritage, régulée par la lapidation médiatique. Oligarchie, car la pratique constante, le Conseil constitutionnel et l'instauration du quinquennat jointe à l'inversion du calendrier électoral ont fait du président de cette république consulaire, à la fois le chef de l'exécutif et celui de la majorité parlementaire, à laquelle il « fixe le cap devant le Congrès. Manque seulement un statut de la « Première dame », ce qui ne saurait tarder. Pas de séparation des pouvoirs donc, sauf pour les constitutionnalistes ayant de bons yeux. La « gouvernance » de cette république s'apparente à une cogestion de la nébuleuse politique présidentielle, de la haute bureaucratie d'État et des fondés de pouvoir des milieux d'affaires- finance et très grandes entreprises. À cette altitude, plus de distinction public-privé. Quel sens pourrait-elle avoir ? La fonction de l'État n'est plus de faire prévaloir un intérêt général, distinct des intérêts particuliers, mais d'assurer la « concurrence libre et non faussée » des acteurs, l'intérêt général résultant du bon fonctionnement du marché, non des équilibres dont l'État est le garant. D'où la porosité de plus en plus grande entre administration publique et direction des banques ou des grandes entreprises privées : pantouflages et rehaussés de passages par les cabinets ministériels ou élyséens. L'explosion des Autorités administratives indépendantes, la diversification des formes de partenariat public-privé, agences de conseil en tout genre adossées à l'État en sont l'expression. Mention spéciale pour les opérateurs de téléphonie mobile et de numérique, régnant par ailleurs sur les médias, dont l'activité et l'enrichissement dépendent de l'autorisation d'exploitation du domaine public par l'État et de la régulation des agences. Les médias sont en effet essentiels à la stabilité du système : propriétés d'une dizaine de milliardaires largement adossés à l'État, ils fabriquent le consensus politique sans lequel il ne saurait se perpétuer. Laurent Mauduit peut même écrire que « jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la liberté et le pluralisme de la presse n'ont à ce point été menacés ; jamais le droit de savoir des citoyens n'a été à ce point malmené. » Ils protègent aussi ce bricolage menacé par une fièvre démocratique endémique en assurant une pression constante sur le seul vestige de pouvoir susceptible de perturber le et cette belle harmonie : le Parlement. Telle est la fonction de la lapidation médiatique qui présente, en outre, l'avantage de faire vendre, pour un investissement intellectuel minimum et sans risque. La manière dont François Fillon a été neutralisé au terme d'une longue carrière politique, traversée sans défrayer la chronique judiciaire,

un peu moins pires que ce qu'ils auraient pu être, mais toujours pas à la hauteur des enjeux. C'est au terme de cette discussion que les membres du RDSE, dans leur diversité, se détermineront. La

les deux projets de loi qui nous réunissent aujourd'hui ont pour principal objet de répondre à un engagement de campagne du Président de la République, inspiré à cet égard par François Bayrou : moraliser la vie publique. C'est un sujet ancien, presque éternel. J'ai relu sur ce point Montesquieu : « C'est

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Trouver la bonne limite, empêcher les abus, tels doivent être nos objectifs, sans pour autant en venir à un autre danger. cultiver l'antiparlementarisme, flatter la dénonciation gratuite des élus de la République serait tout aussi choquant. Oui, la transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus et l'exemplarité de leur comportement, constituent autant d'exigences démocratiques essentielles. Toutefois, vous l'avez rappelé, madame la garde la quasi-totalité des élus exercent leur mandat avec rigueur, abnégation et un grand sens du service public, et il faut le réaffirmer ici. Certes, la campagne électorale de 2017 a été ce qu'elle fut. Sans doute aurait-elle pu être d'une qualité supérieure. Il n'en demeure pas moins que les « affaires », une fois de plus et toujours une fois de trop, ont obstrué le débat public. Cette situation n'est pas neuve. Ces dernières années, on ne compte plus les chroniques relatant les turpitudes de tel ministre en délicatesse avec ses déclarations d'impôts ou de tel autre aux prises avec des comptes à l'étranger. Il ne tient qu'à nous, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, d'y mettre un terme. Rien ne serait pire qu'une énième loi de circonstance ! Au demeurant, le Président de la République nous a communiqué lundi dernier lors de la réunion du Congrès son souhait d'ouvrir le débat sur la modernisation de nos institutions, notamment du Parlement. Nous avons donc une double exigence à respecter : être collectivement à la hauteur du débat que nos concitoyens attendent de nous engager le chantier de la rénovation de nos pratiques institutionnelles. Pour y parvenir, nous devons, au travers de l'examen de ces deux projets de loi, nous poser quatre séries de questions, dont la réponse aura nécessairement une grande importance dans les mois à venir.

Nous avons vu de nombreux collègues députés renoncer à se présenter à un nouveau mandat. L'accélération des parcours politiques pose la question du statut, dans le sens où elle impose une réflexion sur la formation du parlementaire, sa reconversion et, donc, la prévention des conflits d'intérêts pendant l'exercice de son mandat. À cet égard, le mécanisme de déport prévu par le projet de loi ordinaire interpelle. Comment évaluer les critères en fonction desquels un médecin devenu parlementaire serait empêché de siéger à la commission des affaires sociales, sauf à renoncer à son droit de vote ? Faut-il que les anciens avocats cessent de participer à la commission des lois ? Derrière l'aspect provocateur de la question, on comprend la nécessité, madame la garde des sceaux, de définir un juste équilibre permettant à nos institutions de profiter de l'expérience passée acquise par les uns et les autres, tout en luttant, bien évidemment, contre le conflit d'intérêts. Au passage, j'ose une deuxième provocation et un rappel : le meilleur moyen de lutter contre le conflit d'intérêts est de garantir l'attractivité du mandat parlementaire. Le sujet de l'indemnité, même s'il est toujours difficile à aborder publiquement, mérite d'être éclairé. L'indemnité parlementaire- législative, disait-on à l'époque -a été créée par le décret du 5 mars 1848 instituant le suffrage universel. Dans l'esprit des révolutionnaires de 1848, l'indemnité participait de l'abolition du cens, qui concernait aussi les conditions d'éligibilité. Ici, je citerai l'un de nos illustres prédécesseurs sur ces bancs, Georges Clemenceau, sénateur du Var : « Sous la Restauration, vous l'avez déjà deviné, pas d'indemnité. Sous Louis-Philippe, pas d'indemnité. Régime censitaire. Clemenceau affirmait ainsi le caractère démocratique de l'indemnité parlementaire, qui assure aux représentants du peuple leur indépendance face aux pressions de toutes sortes. Par les temps qui courent, il me semble bon de le rappeler L'attractivité du mandat, c'est aussi la considération portée au travail parlementaire, souvent discret, hors du champ des caméras ou des fils d'information. C'est vrai ! Ce sont également les conditions de prise en charge des frais induits par l'exercice du mandat. Je salue, le travail de la commission des lois et de son rapporteur, qui a oeuvré avec la précision et la prudence de l'horloger. Plusieurs collègues auront des propositions à formuler pour nourrir un débat qui nous réunira à plusieurs reprises dans l'année qui vient. Je ne doute pas que nous parviendrons à définir d'ici à la révision constitutionnelle un équilibre satisfaisant sur lequel nous pourrons construire un Parlement avec, certes, moins d'élus, mais une efficacité qui n'en sera que plus grande. Plus que du statut du parlementaire, ces deux textes posent frontalement la question du statut du collaborateur parlementaire. Personne n'en est dupe, ils trouvent leur origine dans l'article d'un hebdomadaire satirique bien connu daté du 26 janvier dernier. Sans doute la pratique dite des « emplois familiaux » a-t-elle été montée en épingle.

Nous aurons des propositions à faire valoir au cours de ce débat pour sortir de cette situation avec humanité et dignité. En deçà de ce problème, il apparaît que les dérives liées au détournement du crédit accordé pour la rémunération des collaborateurs procèdent de ce que ces derniers n'ont pas eu, pendant trop longtemps, d'existence textuelle avérée au-delà de leurs contrats. À cet égard, les assemblées parlementaires ont effectué d'importants progrès ces dernières années. Le régime d'emploi des collaborateurs est désormais inscrit dans notre règlement. Bien évidemment, beaucoup reste à faire. C'est justement dans les interstices de cet édifice en construction que se nichent les voies de ceux, peu nombreux, qui abusent du système. Les présents projets de loi ont le mérite de clarifier ce problème, bien qu'ils n'abordent pas la question dans sa globalité. Aussi prenons date, dès maintenant, pour engager le travail sur le parachèvement du statut de collaborateur parlementaire. Peut-être l'examen des amendements permettra-t-il d'avancer en la matière. J'évoquerai brièvement la question des moyens d'action du parlementaire. Le Parlement du non-cumul ne doit pas conduire à une fracture entre représentation nationale et action locale. Le mandat du parlementaire ne saurait être une mission purement juridique, textuelle L'action politique se nourrit du concret, donc de la relation à l'action locale. À cet égard, la suppression de la réserve parlementaire, certes compréhensible, peut susciter des interrogations. En effet, la réserve demeure le seul moyen d'action locale propre au mandat parlementaire. J'entends par là le seul moyen concret, au-delà de l'influence et de la capacité que peut avoir un parlementaire à interpeller les pouvoirs publics sur les demandes des collectivités.

Nous savons en outre que les finances locales, rigidifiées par la contribution au redressement des finances publiques, ne permettent pas à de nombreuses communes rurales, mais aussi urbaines, de réaliser des projets d'investissements importants tels que des travaux d'accessibilité, la réfection d'un monument ou l'équipement en défibrillateurs. Je salue le travail réalisé par le rapporteur général de la commission des finances et par la commission des lois. Là encore, nous aurons un équilibre à définir en séance pour vous convaincre, madame la garde des sceaux, de sauvegarder un mécanisme de soutien à l'investissement local

Les affaires, encore et toujours, ont conduit de nombreuses banques à considérer les partis politiques comme des débiteurs à risque, tout au moins en termes d'image. d'un immense problème de confiance entre les banques et la vie démocratique. Comme beaucoup d'autres, j'ai pu expérimenter une telle situation, et je crains que le dispositif proposé par le Gouvernement ne soit quelque peu sous-dimensionné. Concernant le médiateur du crédit, permettez-moi de formuler quelques réserves. Quels seront ses moyens d'action ? Comment l'État parviendra-t-il à le doter du capital de confiance nécessaire, dont il aura pour mission d'abonder les partis aux yeux des banques ? Concernant la banque de la démocratie, nous craignons que le dispositif ne soit pas encore arrivé à maturité. En effet, sur le strict plan constitutionnel, il semble impossible que le Conseil constitutionnel, dont vous connaissez les habitudes mieux que nous, madame la garde des valide une habilitation à légiférer par ordonnance dont le champ est fonction d'une enquête conjointe de l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, et de l'IGF, l'Inspection générale des finances, toujours en cours. Une hirondelle ne fait pas le printemps, et deux projets de loi ne suffiront pas à rétablir la confiance de nos concitoyens dans la vie publique. Oui aux dispositions qui concourent à une meilleure régulation de notre vie publique, mais il faut, dans le même temps, doter les parlementaires d'un vrai statut, tout comme leurs collaborateurs, et de moyens d'action. De ce point de vue, vos textes restent, selon nous, au milieu du gué. Madame la garde des sceaux, nos concitoyens n'ont rien à gagner d'un Parlement affaibli. Faire du Parlement une cible serait le symptôme d'une crise démocratique sans doute plus grave encore que la crise de confiance que ces deux textes cherchent à combattre. En disant cela, je ne vous en fais pas le procès. Au contraire, je souhaite que nous indiquions à tous, ensemble, que nous sommes attachés au parlementarisme, qu'il convient de rénover. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tous. Selon moi, nous pouvons, avec ces deux projets de loi, construire les fondations d'un nouvel acte de renforcement du parlementarisme à la française, après la révision du 23 juillet 2008.

J'ai ma petite idée sur ce point : il est possible que cette rupture remonte aux origines même du pouvoir, un peu comme la crise du cinéma date des frères Lumières Vous nous présentez donc ces textes comme les tout premiers du nouveau gouvernement, au nom d'un sacro-saint principe, la transparence. Telle est l'injonction devenue le mot d'ordre de l'époque, au point parfois de rétrécir le débat que cette question appelle. On pourrait gloser à loisir sur ce rêve, cher à André Breton de la « maison de verre », sur cette frontière poreuse entre la vie privée et la liberté individuelle et les exigences nouvelles de la vie publique. Il n'empêche, on doit accepter cette évidence : la transparence est devenue un fait majeur, alimenté par une circulation sans précédent de l'information, pas toujours vérifiée, rendue possible par les nouvelles technologies. De fait, l'esprit public a changé en profondeur concernant les exigences minimales qu'on attend de celles et ceux d'entre nous qui aspirent à devenir des représentants. Quoi que l'on en pense, je suis de ceux qui prennent

quoi qu'en pensent parfois certaines associations spécialisées dans la lutte contre la corruption, nées de manquements constatés ou invoqués à la morale publique. Une partie d'entre elles - pas toutes - versent parfois dans un néo-puritanisme à la scandinave, qui n'est pas, certains le regretteront, dans notre culture politique. Naturellement, quand il est question de morale, on peut tomber dans ce que Nietzsche appelait la « moraline », c'est-à-dire cette petite morale, ivre d'elle-même, déversée par des parangons de vertu qui rivalisent dans la surenchère d'incantations, là où, au contraire, une détermination et une attitude sobre et distanciée paraissent nécessaires pour éviter un bûcher purificateur. C'est sûr ! Voilà deux siècles, Jean-Baptiste Laborde ne craignait-il pas le travers d'une certaine mièvrerie en écrivant : « On aime à blâmer les vices que l'on n'a point, parce que c'est une manière tacite de se louer. » Le Nouveau Testament ne disait pas autre chose : « N'allez pas pratiquer la vertu avec ostentation pour être vu des hommes. » Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs », ajoutait Voltaire. Toute morale, y compris publique, est relative, historique, partielle. C'est la limite du texte qui arrive en discussion aujourd'hui : chacun se croit unique et peut se découvrir quelconque.

l'exemple. Vous pourrez le constater au cours de l'examen des articles, le Sénat a véritablement complété, enrichi et fortifié votre projet, par des propositions sérieuses et neuves comme la création d'un registre des déports pour le Conseil des ministres ou encore la transparence, attendue, des réserves ministérielles.

et avant que l'examen ne s'engage au fond, ce projet comporte des dispositions fort disparates, dont la cohérence d'ensemble n'est pas la première qualité. Extension du régime d'inéligibilité et d'incompatibilités, suppression de la réserve parlementaire, interdiction des emplois familiaux, fixation des conditions de remboursement des frais de mandat des parlementaires et encadrement du financement des partis politiques : il y a là des mesures fort différentes, dont l'efficacité dépendra des modalités de mise en oeuvre. Très franchement,

de discuter du cas de figure singulier et anachronique qui permet encore d'exercer un mandat électif et des fonctions de direction d'un groupe de presse. Ces réserves étant faites, ces textes se révèlent nécessaires, à condition de rappeler que la question morale n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique,

au grand Colbert, dont la statue orne le petit hémicycle et surveille les sénateurs. On sait en effet que le contrôleur général des finances de Louis XIV, grand argentier du roi, n'était pas aussi désintéressé que l'on croit,

». N'a-t-il pas néanmoins sauvé les intérêts majeurs de notre pays au Congrès de Vienne en 1815 ? Je ne cherche pas à jouer du paradoxe. Évitons simplement les mauvais procès en vertu, en surjouant l'indignation. Nous le savons tous, la loi a ses limites. C'est pourquoi il faut avoir à l'esprit

finalement, atrophié le débat de fond qui aurait dû prévaloir dans notre pays, pour choisir le candidat le plus apte à exercer la fonction suprême. De même, j'ai observé l'emballement

D'ailleurs, je note sans malice, madame la garde des sceaux, que le nouveau gouvernement a lui-même pu mesurer cette pente dangereuse fort glissante, si j'en juge par les changements ministériels intervenus précipitamment, qui menacent la stabilité de tous les gouvernants. Défions-nous de ce désir d'un supplément de transparence, qui peut vite se transformer en « tir au pigeon », mû par une certaine jubilation pernicieuse, que je perçois ici ou là dans la presse. C'est une forme de joie mauvaise

pas, ne doit pas nous détourner des enjeux vitaux de notre pays et, donc, de votre capacité à réduire le chômage de masse et la pauvreté que connaît notre pays, à vaincre le terrorisme qui a ensanglanté la France et à annihiler sa menace permanente, à combattre la violence quotidienne, à relever l'école, qui ne remplit plus sa mission première, à enrayer la crise migratoire majeure que subi notre pays et l'Europe et, plus généralement, à sortir de l'impuissance publique généralisée.

tout est immédiatement visible. Le rôle du Parlement et de ses membres doit donc évoluer, pour mieux interagir avec l'ensemble de la société. De ce point de vue, il est regrettable que l'agenda retenu pour l'examen de ce texte, pourtant fondamental pour progresser dans la confiance dans la vie démocratique, n'ait pas permis

aborder la question des licenciements, dans l'esprit dans lequel le président de la commission des lois l'a fait dans son rapport. Concernant les activités de conseil des parlementaires, il faut effectivement mieux déceler et empêcher les conflits d'intérêts. Nous vous suivrons dans cette voie, madame la garde des sceaux,

seront plus touchées par les dispositions prévues que celles qui travaillent dans le secteur public. Il faudra trouver les moyens d'assurer un équilibre, afin qu'il soit

des partis politiques européens. Nous parlons du financement de la vie politique ; il faudra bien, un jour, que nous discutions du financement de la vie politique européenne et de la relation entre les partis politiques européens et les législations nationales. Aujourd'hui, en la

Si ces textes répondent à une profonde attente des Français, certains points méritent cependant réflexion. Pour le moins ! S'agissant tout d'abord de la réserve parlementaire, je me félicite que la commission, si bien présidée-

ne sont parfois éligibles à aucune autre subvention. Si le principe de la réserve parlementaire n'est pas totalement supprimé, le dispositif issu de l'examen du texte par la commission des lois est cependant perfectible. Est ainsi créé le principe d'une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements. Le bénéfice de cette dotation est réservé aux projets d'investissement matériel et immatériel

La liste des projets que les députés et sénateurs souhaitent soutenir sera adressée au Gouvernement par le bureau de chaque assemblée. Le texte est aujourd'hui muet sur les conditions de répartition de la dotation. part minimum de cette dotation doit être garantie à chaque parlementaire pour lui permettre de soutenir son territoire. En l'état du texte, ce minimum n'est pas garanti. pour éviter toute dérive politique, chaque parlementaire doit disposer d'une somme identique. Aucun territoire ne doit être oublié Par ailleurs, je regrette que les associations soient définitivement exclues du bénéfice de ce dispositif. En effet, par exemple, ma région, la grande région

le problème est réel ! Soulignons enfin le « deux poids, deux mesures » du Gouvernement, qui souhaite supprimer la réserve parlementaire tout en conservant les réserves ministérielles. Or, si l'on sait avec certitude que ces dernières sont utilisées à des fins politiques, on ne connaît ni leur montant ni leur destination. En outre, à ces réserves ministérielles s'ajoutent les sommes allouées aux associations sous forme de subventions en 2015, l'État a distribué près de 2,06 milliards d'euros de subventions aux associations, en toute opacité. L'exigence de transparence doit être la même pour tout le monde. S'agissant des incompatibilités, le texte est encore trop imprécis. En l'état, un avocat

On lui demanderait donc de perdre son travail et sa clientèle naissante, alors que l'avocat qui exerce depuis vingt ans, lui, pourrait continuer son activité ! Une telle mesure, qui revient à discriminer la jeunesse, favorisera inévitablement la professionnalisation de la vie politique., politique., sauf erreur de ma part, rien n'empêche le salarié d'une société de lobbying de se présenter aux élections. Le lobbying est une activité de conseil

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, messieurs les rapporteurs de la commission des lois et de la commission des finances, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer sincèrement le travail de fond réalisé en peu de temps par nos collègues des commissions saisies. L'examen de ce projet de loi et de ce projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique est en effet très attendu par nos concitoyens. matière, depuis de nombreuses années, plusieurs textes ont été adoptés- notre collègue Jean-Pierre Sueur a évoqué quelques dates, dont certaines sont lointaines. S'agissant de la transparence, la mise en place de la Haute Autorité

nationaux, nous nous devons de rendre des comptes. L'éthique, la morale, la transparence, l'exemplarité, sont des priorités. D'où l'importance des hautes juridictions, telles que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, et des tribunaux administratifs. Depuis plusieurs années, sur l'initiative

Nous sommes responsables de l'argent public ; élus, nous le sommes pour servir l'intérêt général. Le dévouement des élus locaux et nationaux mérite d'ailleurs d'être souligné, et je vous remercie, madame la garde des sceaux, de votre témoignage en ce sens.

serait très regrettable, d'autant plus que son utilisation, dans le cadre de la dotation d'action parlementaire, est parfaitement encadrée.

L'instruction de ces dossiers par le ministère de l'intérieur est totalement transparente : devis estimatif et quantitatif, attestation de non-commencement des travaux, plan de financement, etc. Les notifications de subventions signées par les ministres de l'intérieur successifs

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, merci infiniment de vos interventions, que j'ai trouvées extrêmement riches, bien qu'elles aient parfois été critiques.

Il me semble que, parmi les éléments de réponse que j'apporterai et dont nous discuterons dès demain, ce souci de convergence apparaît, puisque le Gouvernement a d'ores et déjà entendu un certain nombre de préoccupations que vous avez exprimées sur la limitation de l'indemnité perçue par les ministres quittant leur fonction, sur l'attestation fiscale

parlementaires membres de la famille d'un parlementaire aient le temps de se retourner- nous y reviendrons également. Le Gouvernement a donc d'ores et déjà pris en compte un certain nombre de vos

une institution suffisante pour remédier à l'ensemble des difficultés rencontrées par les partis politiques ou les candidats à une élection. C'est pour cette

souhaite également que soit mis en place, si je ne déforme pas ses propos, un statut plus général pour les collaborateurs parlementaires. C'est une question qui a été reprise également par d'autres sénateurs.

Du fric-frac au ping-pong, je suis certaine que nous arriverons à trouver un accord sur ce point ! Vous avez encore évoqué la question de la limitation des activités de conseil.